Mes chers collègues, pour le respect des règles sanitaires, je vous rappelle qu'il convient de laisser un siège vide entre deux sièges occupés ou, à défaut, de porter un masque. Je vous rappelle également que les sorties de la salle des séances devront exclusivement s'effectuer par les portes situées au pourtour de l'hémicycle.

objet : la création d'un fonds d'urgence de 10 millions d'euros pour les ressourceries et recycleries. Cette question a déjà été abordée à l'Assemblée nationale, et nous n'avons pas été totalement rassurés quant à la volonté de soutenir les structures de l'économie sociale et solidaire (ESS), qui relèvent Merci Quelques mois après le vote de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, et alors que les Français sont de plus en plus attachés au développement d'une société plus vertueuse, il paraît indispensable de venir en aide à ce secteur.

serait destiné aux associations, comme Emmaüs, qui, pour la première fois de son histoire, en a appelé à la générosité, faute de dons. Le fonds Itier n'est pas opérant dans ce cas précis. Notre demande est donc claire : il faut présenter la mise en place d'un fonds d'urgence pour l'économie sociale et solidaire lors d'un conseil d'administration extraordinaire de l'Ademe. Dans cette attente, M. Bigot souligne le caractère indispensable de cet amendement pour les ressourceries et recycleries.

L'ensemble des structures de spectacle vivant, les diverses industries culturelles, tous les contributeurs à la création et le secteur du patrimoine se trouvent dans des situations très difficiles. Tous ces acteurs ont pâti de l'annulation des manifestations culturelles et artistiques, de la fermeture des musées, monuments, salles et lieux de pratique culturelle ; et les industries culturelles ont subi les dommages collatéraux de ces fermetures et annulations. Pour l'heure, nous considérons que la culture n'a fait l'objet d'aucun plan d'envergure, contrairement au secteur du tourisme : elle n'a bénéficié que de simples mesures sectorielles, qui, pour nous, relèvent davantage du saupoudrage. Nous proposons donc un fonds doté de 2 milliards d'euros pour financer : un fonds de soutien au spectacle vivant ; un fonds de soutien aux artistes et techniciens du spectacle vivant ; la modernisation des salles de spectacle- ces dernières pourraient ainsi investir dans du matériel de captation audio

; un fonds de soutien aux artistes plasticiens et visuels ; un élargissement du périmètre du fonds pour l'emploi pérenne dans le spectacle ; un abondement exceptionnel du fonds de soutien à l'expression radiophonique ; un fonds d'urgence pour la presse indépendante ; enfin, un fonds d'urgence pour le patrimoine.

et la période de confinement que nous venons de vivre rappellent combien la question de l'accessibilité et de la médiation numérique est essentielle pour la cohésion sociale de notre pays. La fracture numérique entraîne une rupture d'égalité inacceptable entre les citoyens, accentuant les situations de détresse, d'isolement et de précarité des personnes qui sont coupées du numérique. L'équipement des foyers en matériel informatique s'est également révélé être un facteur supplémentaire de rupture d'égalité faire l'école à la maison est vite devenu un défi insurmontable pour de nombreuses familles. Le redressement de la France doit passer par un égal accès de tous à un internet de qualité et par une véritable appropriation par les citoyens du numérique et de ses usages. Malgré les actions menées depuis une

La responsabilité de l'État est d'agir pour aider à réduire les fractures induites par les évolutions technologiques et sociétales. Cette action passe par le déploiement de moyens massifs pour accompagner les publics les plus éloignés du numérique. Il est nécessaire de construire une stratégie numérique républicaine englobant les infrastructures, les services et les usages, pour un numérique durable au service de tous nos concitoyens. Cet objectif d'inclusion sociale doit être placé au coeur de la relance de notre pays.

Ce fonds sera fléché vers les outils d'accompagnement mis en place par les régions ou par les professions, quand celles-ci disposent d'une structure de capital-risque. Les comités professionnels de développement économique, le DEFI et Francéclat ont aussi été particulièrement touchés. Ils ont

en faveur des entreprises exerçant leur activité dans les collectivités ultramarines afin de leur permettre de bénéficier d'une aide budgétaire exceptionnelle en compensation des surcoûts engendrés par la crise de la covid.

les mesures de recours à l'activité partielle n'ont pas pu s'appliquer aux entreprises exerçant leurs activités dans les collectivités ultramarines du Pacifique. Il est donc proposé de créer une aide budgétaire exceptionnelle d'urgence visant à prendre en charge ces surcoûts pour les entreprises des secteurs les plus touchés et dont certains, comme le BTP,

d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action n° 01, Favoriser le recours à l'activité partielle pour prévenir les licenciements, du programme 156 et à ouvrir, en contrepartie, 150 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sur l'action n° 01, Fonds d'urgence pour les entreprises des collectivités ultramarines,

des garanties données par l'État et passer à des aides budgétaires, c'est-à-dire à des subventions. Les régions font ce qu'elles peuvent, mais ce n'est pas véritablement opérant. Nous demandons donc au Sénat et au Gouvernement de comprendre ces problèmes structurels

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). On sait que le droit commun pose souvent problème. J'entends notre excellent rapporteur général évoquer le dispositif de l'AFD.

demandons la création d'un fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection des réseaux d'eau en Guadeloupe. Sur « l'île aux belles

accru la probabilité de contamination, de morbidité, voire de mortalité en Guadeloupe. Le Président de la République s'est engagé à octroyer, tenez-vous

», dotée de 4,5 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Les médias généralistes privés d'outre-mer jouent un rôle indispensable à la pluralité de l'information dans les territoires dans lesquels ils sont implantés. Ils occupent souvent une position de leader d'audience et rassemblent quotidiennement 1,5 million de téléspectateurs et d'auditeurs en Martinique, en Guadeloupe, à la Réunion et en Polynésie,

Pendant le confinement, ces entreprises ont poursuivi leurs missions d'information et de divertissement de la population, engageant des frais supplémentaires pour couvrir l'évolution de la situation sanitaire. Elles n'ont pas pu bénéficier des aides d'urgence mises en place par l'État, telles que l'activité partielle et le fonds de solidarité, alors qu'elles faisaient face à un effondrement face à un effondrement de 90 % de leurs recettes, et se trouvent aujourd'hui dans une situation extrêmement préoccupante, qui met en péril la pérennité de l'emploi et l'existence même de certaines d'entre elles.

La crise sanitaire a eu un impact important sur les enseignants-chercheurs non titulaires de l'enseignement supérieur, entravant largement l'avancée de leur thèse. Sans prolongation systématique de leur contrat de travail, ces jeunes scientifiques et leurs projets, dont beaucoup sont en lien avec les crises climatiques, écologiques, sanitaires, sociales ou économiques actuellement éclipsées par la covid-19, seront des victimes collatérales de l'épidémie

Toutefois, les annonces de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le financement de cette prolongation des contrats doctoraux ont été suivies d'un grand flou et les principaux intéressés se sont trouvés confrontés au silence de leurs administrations démunies. N'ayant pas pu, pour le moment, obtenir de rallonge budgétaire suffisante pour financer cette mesure, plusieurs directions de recherche ont adressé aux directrices et directeurs de laboratoires des instructions pour procéder à une sélection des doctorants qui pourront en bénéficier. Faute de Faute de financements suffisants, l'annonce ministérielle contraint ainsi nos universités à procéder à des sélections sur des critères établis en toute hâte. La situation est donc très préoccupante et risque de concerner beaucoup de doctorants

villages à offrir des services au titre de leur rôle de centralité, mais également à soutenir des villages qui, dans le cadre d'un maillage particulier, remplissent des fonctions indispensables à la population

Toutefois, alors que la saison estivale a commencé, aucun dispositif opérationnel d'urgence n'a été mis en place. Faut-il rappeler qu'une étude récente réalisée par la fondation Jean-Jaurès et l'IFOP révélait que deux tiers des Français avaient été contraints de renoncer à partir en vacances d'été pour des raisons financières traversons ne peut qu'aggraver cette situation alors qu'un soutien fort de l'État aux départs en vacances et aux structures du secteur était attendu. La crise frappe les ménages déjà pauvres, mais aussi ceux qui ont des revenus intermédiaires, car plus d'un tiers des actifs ont vu leurs revenus d'activité baisser. Les secteurs du tourisme social et solidaire les plus fragilisés sont les organisateurs de colonies de vacances et de vacances adaptées aux personnes en situation de handicap. Le nombre d'enfants ou de jeunes accueillis cet été est en forte baisse, car des séjours ont été annulés ou la capacité d'accueil des structures a été réduite.

Pour favoriser des vacances pour tous, il était pourtant urgent de déployer une communication et des aides massives de manière à susciter la demande et à sécuriser l'offre, avec un soutien rapide au secteur du tourisme social et solidaire. Les sénateurs du groupe socialiste et républicain ont déposé, le 15 mai dernier, une proposition de loi favorisant des vacances pour tous cet été, avec deux dispositifs : un chèque-vacances « Solidarité 2020 » à destination des familles modestes, financé par l'État et les collectivités territoriales ; un soutien d'urgence au tourisme social et solidaire et aux organismes de colonies de vacances s'inscrivant dans le cadre d'un tourisme durable et de proximité, afin qu'ils soient en mesure de proposer une offre adaptée

le bénéfice de ce fonds, aux mêmes conditions, aux entreprises de certains secteurs qui dépendent fortement de ceux que je viens de citer et qui ont perdu plus de 80 % de leur chiffre d'affaires entre le 15 mars et le 15 mai En conséquence, à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a doté le fonds de 500 millions d'euros supplémentaires. Pour autant, ce fonds continue de souffrir d'un certain nombre de lacunes, qui nuisent à son efficacité. D'une part, l'assouplissement des critères d'éligibilité s'applique

cet assouplissement des critères n'est effectif qu'en cas de baisse du chiffre d'affaires de 80 % durant les deux mois de confinement. En conséquence, une entreprise ayant subi une baisse de 75 % de son chiffre d'affaires est exclue de ce dispositif spécifique. Notre cellule « PME, commerce et artisanat » salue l'assouplissement déjà réalisé des critères d'éligibilité,

au Gouvernement de pérenniser le fonds de solidarité jusqu'à la fin de l'année, et surtout de renoncer à une logique de soutien sectoriel en optant pour une logique fondée sur les difficultés réelles des entreprises.

retrait, monsieur le rapporteur général,

pour surmonter les effets de la crise sanitaire, les entreprises qui emploient des intermittents du spectacle ont été particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la pandémie de covid-19.

qu'un très grand nombre d'employeurs éprouvent des difficultés à assumer le règlement de ces cotisations sur l'indemnité d'activité partielle, la caisse pourrait ne plus pouvoir procéder au paiement des indemnités

amendement vise à abonder la ligne budgétaire de prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel faisant suite à la crise sanitaire, afin d'accompagner ces entreprises dans le paiement des cotisations dues à la caisse des congés spectacles.

Je confirme l'analyse, en ajoutant que le dispositif proposé par Mme la sénatrice nous paraît redondant avec le maintien des droits acté jusqu'au 31 août 2021. Avis défavorable. Madame Dumas,

Au sein de la mission « Recherche et enseignement supérieur », le présent amendement vise à annuler 600 millions d'euros de crédits pour le programme « Recherche spatiale » pour ouvrir 300

à soutenir l'économie et les entreprises. Pourtant, la crise sanitaire a eu d'importantes conséquences sur d'autres pans de notre société, à commencer par l'enseignement supérieur. Ainsi, certains étudiants, démunis d'outils numériques, n'ont pu suivre l'ensemble des cours, ni accéder aux bases de données des universités, ni échanger avec les enseignants

De plus, les étudiants les plus précaires ont été durement touchés par la crise sanitaire, et cette situation risque de perdurer, certains ayant du mal à trouver un emploi pour l'été. C'est pourquoi il convient d'aider ces étudiants en augmentant les bourses qui leur sont destinées.

de la recherche publique, notamment de ses deux grands opérateurs, le CNRS et l'Inserm. Mes chers collègues, il faut que vous compreniez bien dans quelle situation paradoxale se trouve la recherche française. Nos collègues

Alors que nos citoyens demandent à la science de leur proposer demain, pour sortir de cette pandémie, des solutions thérapeutiques et un vaccin, notre pays n'investit pas dans cette recherche.

heures 43 sur une radio nationale, que l'investissement dans la recherche est une nécessité absolue, pourquoi ne pas commencer en 2020, année de la pandémie ?

urgente au déficit majeur de financement public de la recherche médicale. C'est maintenant qu'il faut le faire ! Il est incompréhensible que l'Allemagne investisse à hauteur de 4 milliards

dans une position défavorable pour la négociation de l'achat du futur vaccin, car je peux vous assurer que Sanofi ira au plus offrant, c'est-à-dire vers l'Allemagne, qui met 4 milliards d'euros ou vers les États-Unis, mais pas vers la France qui en met zéro. Vous envoyez un message extrêmement négatif

On parle beaucoup de santé personnalisée et de traitements innovants : donnons aux chercheurs les moyens de trouver de nouveaux traitements intéressants.

directes, du programme 231, « Vie étudiante », finance des aides directes pour les étudiants. Dans ce cadre, la loi de finances pour 2020 a prévu de transférer 4 millions d'euros à Bpifrance afin de financer son fonds de garantie « Prêts Étudiants Ce dispositif a un effet de levier important puisque, en 2019, quelque 3 000 étudiants ont ainsi pu obtenir un prêt garanti à 70 % par l'État pour un total de 24 millions de prêts, soit une moyenne de 8 000 euros par prêt. L'enveloppe augmentée pour 2020 à 4 millions d'euros reste insuffisante, puisque Bpifrance réclamait 5,5 millions d'euros de crédits annuels afin d'atteindre un montant total de 100 millions d'euros de prêts. Cela permettrait aux banques de commercialiser ce produit plus largement et plus longtemps. L'enveloppe est d'autant plus insuffisante cette année que les conséquences économiques de la crise que nous traversons laisseront inévitablement des traces dans le budget des familles les plus modestes. Or, comme le disait notre collègue Pierre Ouzoulias,

nous avons bien mentionné que le milliard d'euros supplémentaires feraient l'objet d'un report de crédits si les travaux n'étaient pas engagés aussi rapidement que d'habitude. La parole

durable, dite Égalim, a constitué une véritable avancée puisqu'elle a fixé des objectifs d'au moins 50 % de produits sous signe de qualité et de 20 % de produits bio d'ici à 2022, les restaurants collectifs restent encore aujourd'hui loin du compte, avec, notamment, seulement 4,5 % de bio servi selon l'Agence Bio. S'il est possible d'atteindre ces objectifs sans surcoût final comme l'ont montré de nombreux exemples locaux, pour lesquels,, le prix à l'assiette était identique, la transition nécessite temporairement des moyens, notamment pour construire et structurer des circuits d'approvisionnement locaux en lien avec les acteurs du territoire, sensibiliser les usagers, former les personnels, ou encore réaliser des diagnostics, notamment

de produits frais. Cet amendement vise donc à financer ce surcoût temporaire, qui permet l'enclenchement d'une boucle vertueuse, puisque la réduction du gaspillage et le travail de produits bruts, locaux, de saison, les restaurants réalisent des économies qu'ils peuvent ainsi réinjecter dans l'achat de produits bio et de qualité. Nous proposons de créer un programme Aide à la transition alimentaire de la restauration collective publique », doté de 15 millions d'euros, afin de soutenir les collectivités locales dans la transition alimentaire de la restauration collective publique.

rémunérés à un prix juste. Cette recherche d'équité se doit d'être renforcée à l'heure de la crise sanitaire, économique et sociale que nous vivons. De plus, financer l'atteinte des objectifs de la loi Égalim est un levier pour développer notre souveraineté alimentaire,

de véhicules pour la police, pour un montant de 60 millions d'euros en crédits de paiement : 1 150 véhicules à motorisation essence, 1 150 véhicules électriques, mais aussi 1 500 vélos électriques dans les zones les plus urbaines. Quel est l'avis

de réduire autant la flotte des véhicules, tant de la police que de la gendarmerie. Cela conduit évidemment nos forces de l'ordre à courir derrière des voleurs qui, eux, roulent en 4x4 surpuissants

qui bénéficient aujourd'hui de cette aide. L'amendement reprend l'une des propositions du plan de rebond économique, social, écologique présenté par le parti socialiste le 9 juin dernier, qui tend à créer un fonds de soutien de 100 millions d'euros à destination des associations d'aide alimentaire. Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il était nécessaire de le gager. En conséquence, nous proposons de diminuer respectivement de 45 millions et de 55 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement le budget des actions n 11 et 12 du programme 124, et d'augmenter de 100 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement celui de l'action n° 14 du programme 304. Quel est l'avis de la commission ?

navette. Quel est l'avis de la commission ?

retrait, monsieur le rapporteur général,

L'amendement vise à aligner les dispositifs des contrats de professionnalisation sur les dispositifs d'apprentissage en matière d'octroi de la prime exceptionnelle d'embauche des apprentis.

par le Gouvernement. Il y avait un autre calendrier possible ! Je vous rappelle que le Président de la République a souhaité que son Premier ministre s'exprimât

M. le ministre délégué. La question que pose M. Ouzoulias relève du champ réglementaire, je le précise. À ce stade, et de mémoire, parce que je ne l'ai pas vérifié à l'instant, le dispositif d'aide à l'apprentissage ne couvre pas les formations de niveau master et au-delà.

de ce secteur permettrait de compenser partiellement les pertes de chiffre d'affaires et d'exploitation des entreprises concernées et de couvrir les surcoûts liés au maintien d'activité et à la poursuite des actions d'accompagnement à distance des salariés en parcours d'insertion.

une partie de nos jeunes et induit une perte de compétences intolérable, l'aide restant conditionnée à l'apprentissage et n'étant pas ouverte aux primo-accédants

Monsieur le ministre, nous savons tous que la rentrée sera violente sur le marché de l'emploi, notamment pour les jeunes ; je n'imagine pas que vous ne soyez pas favorable à cette mesure

appelons le Gouvernement à modifier les conditions d'attribution de la prime exceptionnelle à l'embauche d'apprentis. Cette prime concernerait les apprentis visant l'acquisition d'un diplôme allant du CAP à la licence professionnelle. Fixée à 5 000 euros pour les apprentis mineurs et à 8 000 euros pour les apprentis majeurs, selon les annonces du Gouvernement, elle serait versée sans condition aux entreprises de moins de 250 salariés. pour les entreprises de plus de 250 salariés, le Gouvernement conditionnerait son octroi à un objectif de 5 % d'apprentis dans l'effectif total de l'entreprise. À défaut, l'aide devrait être remboursée. Ce seuil minimal nous paraît dissuasif et de nature à freiner l'embauche d'apprentis, car de nombreuses entreprises sont bien en deçà de ce seuil. En second lieu, cet amendement vise à mieux soutenir l'embauche d'apprentis par les entreprises, en complétant l'aide à l'embauche annoncée par le Gouvernement le 4 juin 2020. Il est notamment nécessaire que cette aide soit allouée quel que soit le niveau de diplôme préparé, plutôt que de la limiter aux formations jusqu'au niveau licence, afin de ne pas introduire de rupture d'égalité entre les apprentis.

Comme le souligne ce rapport, l'urgence est, aujourd'hui, de prévoir les mesures qui éviteront de faire de l'apprentissage l'une des premières victimes de la crise économique. Alors que ce mode de formation était à nouveau en progression, la tendance risque de connaître un coup d'arrêt brutal. Le contexte actuel justifie pleinement que le Gouvernement s'engage à prendre de telles mesures.

venir financer une partie de l'apprentissage effectué dans la fonction publique. Ce décret d'application a également été accompagné d'un arrêté prévoyant que, si jamais les crédits demandés au CNFPT excédaient 25 millions d'euros, France compétences viendrait en relais.

prévoyant notamment une avance de l'Agence France Trésor d'un montant de 100 millions d'euros au bénéfice du réseau de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE), qui a particulièrement souffert de la crise sanitaire et économique. Interpellé par plusieurs d'entre nous, le Gouvernement s'est par la suite engagé, au cours d'une audition, à transformer cette avance en crédits ou dotations. ou dotations. Il n'a qu'à moitié respecté sa parole, puisque 50 millions d'euros ont effectivement été crédités sur le programme 185, « Diplomatie culturelle et d'influence », de la mission « Action extérieure de l'État », tandis que 50 millions d'euros sont toujours crédités sous la forme d'avance sur le programme 823, Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics ». Au-delà des promesses gouvernementales, qui n'engagent que ceux qui les croient, il me semble essentiel que ces 50 millions d'euros d'avance soient crédités directement sur le programme 185 de la mission « Action extérieure de l'État En effet, il est certain que le remboursement de cette avance sera supporté par les familles du réseau AEFE sous la forme d'une nouvelle hausse des frais de scolarité. Ces familles sont pourtant déjà lourdement mises à contribution puisqu'elles participent à hauteur de 70 % au financement du réseau et que cette proportion ne cesse d'augmenter au fil des ans. Le maintien de cette avance de 50 millions d'euros, qui devra être remboursée dans un délai utopique d'un an, révèle encore une fois le désengagement progressif de l'État dans l'AEFE, un outil pourtant essentiel de la diplomatie culturelle française dans le monde. Un amendement de transfert de crédits entre deux missions étant considéré comme irrecevable, je demande une nouvelle fois au Gouvernement de bien vouloir transformer cette avance de 50 millions d'euros en crédits,